Dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane, cet amendement vise à créer une infraction de détention et de transport non justifié d'une grande quantité de carburant. En effet, le carburant est le nerf de la guerre.

ne conduisent qu'à très peu de bassins de vie justifiant l'acheminement de carburant en très grande quantité. L'essentiel du carburant qui transite sur ces cours d'eau est destiné à l'orpaillage, parfois légal- auquel cas le transport de carburant est justifié -, mais souvent illégal. proposons donc de créer une infraction permettant de saisir le carburant avant même que celui-ci ne soit livré à un site d'orpaillage illégal et de poursuivre le détenteur ou le transporteur, dans le but de juguler les trafics qui approvisionnent les exploitants clandestins. Quel

Ce dispositif permet d'accentuer la lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane, dans la mesure où le transport d'une grande quantité de carburant peut être vu comme l'indice d'une activité illégale d'extraction. La commission

sans être en mesure de fournir la référence du permis, de l'autorisation ou du titre minier dans lequel ce matériel est destiné à être utilisé, mais aussi à confisquer le matériel en question. l'amendement vise à punir de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait, dans le cadre d'une activité d'orpaillage illégal, de charger, de décharger ou de transborder un bateau, un engin flottant, un matériel flottant ou un véhicule terrestre à moteur.

vise à introduire un nouveau facteur aggravant de la sanction pénale pour l'exploitation de mine sans titre dans les espaces naturels protégés. En effet, si le code minier prévoit actuellement une aggravation de la peine pour les infractions d'exploitation de mine sans titre, en raison du rejet ou du déversement de substances nocives pour la santé ou à l'environnement, de l'émission de substances constitutives d'une pollution atmosphérique, de la coupe de bois ou de forêts, de la production ou de la détention de déchets dans des conditions de nature à porter atteinte à la santé et à l'environnement, il ne traite pas de la question de l'exploitation de mine sans titre dans les espaces naturels protégés. Or l'orpaillage illégal touche de plus en plus les zones faisant l'objet de mesures de protection du patrimoine naturel, en particulier le parc amazonien de Guyane ;

C'est pourquoi nous proposons d'ajouter à la liste des facteurs d'aggravation de la peine encourue en cas d'exploitation de mine illégale, le fait de prospecter sans titre dans un espace naturel protégé, ce qui permettra d'augmenter l'exemplarité de la sanction pénale et de renforcer la cohérence de la lutte contre l'orpaillage illégal

Deuxièmement, l'effet dissuasif d'une interdiction du territoire français n'est absolument pas prouvé. La frontière guyanaise est d'abord une rivière, puis une jungle, difficile si ce n'est impossible à surveiller. En outre, on s'adresse à des personnes qui, vraisemblablement, traversent les frontières plusieurs fois par jour sans se soucier de savoir si le territoire français leur est interdit ou non. Troisièmement, cet article va à l'encontre va à l'encontre du droit d'asile. Or la région entourant la Guyane n'est pas à l'abri de déstabilisations politiques profondes, comme nous le voyons au Brésil, en Colombie et au Venezuela. Cet article signifie donc qu'un individu reconnu coupable d'orpaillage illégal et dont la situation changerait gravement dans son pays d'origine ne pourrait pas demander l'asile en France parce qu'il serait frappé d'une interdiction du territoire français. telle disposition semble en outre aller à l'encontre du principe de non-refoulement issu de la convention de Genève de 1951 et de toutes les dispositions légales nationales relatives au droit d'asile à la frontière, que la France, au-delà de ce délit, doit respecter. Toutes ces contradictions juridiques rendent cet article difficilement applicable, voire « illégal ». C'est pourquoi nous vous en proposons la suppression, sans que cela altère et atteigne par ailleurs les dispositions pénales renforcées déjà prévues en amont de ce texte, que nous approuvons.

162-1 du code minier, ce qui conviendrait au Gouvernement, mais, en réalité, votre rédaction renvoie à l'article L. 162-1 du code de l'environnement. Par conséquent, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur cet amendement, qui ne permet pas au dispositif initialement envisagé d'être opérant sur le fond.

afin d'instaurer un mécanisme de prévention et de responsabilité objective pour les activités d'exploration et d'exploitation des mines. Par cette transposition, les dommages causés à l'environnement par les exploitants pourront être plus efficacement jugés et dédommagés. Quel de la commission ? Cet amendement est pleinement satisfait par l'article 20 du présent projet de loi, introduit en séance à l'Assemblée nationale. Il intègre les activités régies par le code minier dans le champ de la responsabilité environnementale. La commission l'a validé avec plusieurs précisions. La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle

Cet amendement vise à clarifier les délais de transmission à l'autorité administrative de l'étude de faisabilité, au regard du contexte géologique, à l'arrêt effectif des travaux et non seulement à la déclaration de l'arrêt. est de garantir une meilleure sécurité lors des travaux de recherche et d'exploitation de géothermie. La parole l'amendement n° 1835. Le présent amendement a pour objet d'étendre la possibilité, pour l'autorité administrative, de demander aux exploitants d'installations géothermiques existantes la production et l'actualisation d'un mémoire sur le risque de sismicité. Cette faculté serait ainsi autorisée jusqu'à l'arrêt des travaux, dans un souci de prévention des risques.

du matériel spécifiquement destiné à l'exploitation aurifère sans être en mesure de fournir la référence du permis, de l'autorisation ou du titre minier dans lequel ce matériel est destiné à être utilisé. Quel est l'avis de la commission des affaires économiques ? L'évolution proposée permet d'instituer une nouvelle infraction, dans le cadre des pouvoirs de contrôle, de vérification ou de relevé d'identité confiés aux officiers de police judiciaire. Cette infraction pénaliserait davantage le transport fluvial non autorisé de matériel utilisé pour l'exploitation aurifère et concourrait à conforter le volet du texte lié à la répression de l'orpaillage illégal en Guyane. La commission émet

Mme Raymonde Poncet Monge. Partout dans le monde, l'extraction de l'or se révèle destructrice pour l'environnement. Une mine d'or est d'abord une usine chimique au milieu de la nature,

et sont parfois déversées volontairement dans les océans, quand ce ne sont pas les cuves qui débordent en pleine forêt amazonienne, comme ce fut le cas de nombreuses fois. L'extraction aurifère industrielle nécessite, par ailleurs, des quantités astronomiques d'eau. En moyenne, 140 000 litres d'eau par heure sont nécessaires, ce qui correspond à la consommation d'eau annuelle d'un foyer de trois personnes en Allemagne. À cela s'ajoute l'abattage d'arbres géants dans les forêts vierges : des pelleteuses creusent la terre, laissant derrière elles des paysages lunaires. En outre, 1 000 kilogrammes de déchets toxiques et de déblais sont produits pour obtenir seulement 0,24 gramme d'or.

En Guyane, les projets de recherches se multiplient, au détriment de la protection de la biodiversité exceptionnelle de ce territoire, et sans que la rentabilité des projets- je ne parle pas de rentabilité privée -soit toujours au rendez-vous.

d'euros de subvention publique, pour seulement douze ans d'exploitation, laissant derrière lui un territoire déboisé et pollué pour plusieurs décennies. À lui seul, il aurait représenté une augmentation d'environ 50 % de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre de la Guyane.

Cet amendement vise donc à proposer un moratoire sur l'exploitation minière industrielle aurifère en Guyane, en vue d'entamer les mesures nécessaires à son interdiction sur le territoire français, comme le réclamait la Convention citoyenne pour le climat. Quel est l'avis de la commission des affaires

de production entre l'une et l'autre. Ensuite, le projet de loi apporte des modifications importantes pour minimiser l'impact de l'exploitation industrielle aurifère, en particulier en Guyane. Enfin, au cours des auditions que j'ai pu réaliser, aucun élu local guyanais n'a émis le souhait d'interdire toute exploitation aurifère. Je veux ajouter, pour conclure, que viser l'ensemble des collectivités ultramarines dans le cadre de ce moratoire serait peu adapté, car seule la Guyane dispose de gisements aurifères. La commission demande le retrait de cet amendement

singulier en matière d'exploitation minière, en raison de la richesse des gisements aurifères qui y sont présents et de l'activité structurante qui en découle. La filière aurifère est ainsi le deuxième secteur industriel du département, après l'aérospatiale, et représente 40 TPE et 5 PME, pour environ 600 emplois directs. C'est pourquoi le Gouvernement a lancé une mission d'inspection afin d'étudier l'avenir de cette filière et de déterminer les engagements volontaires qui permettraient d'en faire une filière pleinement responsable sur le plan environnemental.

Il reste évident- mes collègues l'ont indiqué -que l'orpaillage, particulièrement non régulé, entraîne de nombreuses conséquences négatives pour l'environnement et pour l'être humain, c'est-à-dire pour les sociétés locales.

L'extraction d'une tonne d'or nécessite 150 tonnes de cyanure en moyenne ; en outre, il est parfois fait utilisation du mercure. Cyanure et mercure contaminent les sols et les nappes phréatiques à jamais. ailleurs, les populations autochtones vivant au bord des fleuves, particulièrement exposées à ces produits toxiques, en subissent directement les conséquences. Ainsi, selon l'Institut de veille sanitaire,

cheveu, le seuil tolérable fixé par l'OMS étant de 10 microgrammes. Il revient donc au Gouvernement de rendre au Parlement un rapport sur l'impact économique, sanitaire et environnemental de l'orpaillage en Guyane française, afin de mettre en place une politique plus respectueuse de l'environnement et de mettre en lumière les conséquences sanitaires que subissent les populations concernées, notamment à des fins d'indemnisation, pour ce qui constitue, à tout une imprudence de la part de la puissance publique et, au pire, un crime d'écocide. Quel la commission des affaires économiques n'est pas favorable aux demandes de rapport. Par ailleurs, les sujets soulevés ont vocation à être débattus dans le cadre de la préparation de l'habilitation à légiférer par ordonnances, à laquelle notre commission a

? Madame la sénatrice, la concentration de mercure dans les cheveux ou dans les organismes des populations amérindienne

certains aspects de la fiscalité minière. La fiscalité minière française repose actuellement sur trois redevances au profit des collectivités locales : la redevance communale des mines, dont parlait M. Jacquin, la redevance départementale des mines et la taxe spéciale sur l'or, applicable Le Gouvernement est convaincu qu'il convient de faire évoluer cette fiscalité, afin que celle-ci puisse être mieux répartie au profit des communes concernées par les activités minières. Ce qui a été adopté en commission n'a pas fait l'objet d'une concertation avec les communes concernées. Les sommes en jeu ne sont pas énormes,

Nous devons donc légiférer sur ce point et rapidement. Il ne faudrait pas que la reconquête de notre souveraineté minière ne bénéficie pas, faute d'une fiscalité inadaptée, aux collectivités territoriales. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

le rééquilibrage du produit de la redevance communale des mines concerne les substances minérales et non les hydrocarbures liquides ou gazeux, dont l'extraction est en voie d'extinction sur le territoire national d'ici à 2040, en application de la loi du 30 décembre 2017

initiative, par ordonnance. Madame la ministre, plus que jamais, il faut écouter les maires, les élus des territoires et les citoyens, qui doivent participer aux travaux menant à une réforme en profondeur du code minier.

Cette dernière doit être menée ici, par les parlementaires, après avoir entendu les citoyens et les élus de nos circonscriptions et après avoir constaté,, ce que l'après-mine signifie.

aux ordonnances. L'article 21 est constitué d'une série de déclarations d'intentions du Gouvernement sur lesquelles nous n'avons aucune prise, alors même que la réforme du code minier est un enjeu écologique et stratégique fondamental. Pouvons-nous

par respect pour la démocratie et pour le Parlement et parce que nous voulons une réelle discussion sur un enjeu écologique et stratégique important, nous demandons la suppression de l'article 21, qui habilite le Gouvernement de légiférer par ordonnances.

de gestion des risques miniers résiduels. J'appelle votre attention sur la mobilisation des associations, dont certaines sont bien connues comme l'Association des communes minières et, plus localement, chez moi, en Meurthe-et-Moselle, l'association SEL'idaire ou l'Association des communes du bassin minier

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

d'articulation entre la partie réglementaire du code minier et le code de l'environnement et de consultation d'un large panel représentatif de parties prenantes. Pour aboutir à des textes de qualité permettant de mettre un terme cette réforme du code minier dans les meilleures conditions de concertation, le délai de douze mois ne paraît pas suffisant.

le système d'indemnisation et de réparation des dommages miniers. En effet, le système actuel a largement démontré ses limites, plaçant certains administrés en situation de précarité. L'amélioration du système d'indemnisation est la première des préoccupations des collectivités et de leur population. Aussi, il paraît indispensable que les associations d'élus locaux, les représentants des professionnels et du personnel du secteur minier ainsi que les associations de protection de l'environnement soient consultés sur les décrets d'application relatifs au système d'indemnisation et de réparation des dommages miniers. Quel est l'avis de la commission

les modalités de fonctionnement de cette plateforme, qui permettra de dématérialiser certaines procédures liées à la gestion des titres. Cet amendement tend en outre à élargir l'habilitation à de nouvelles mesures consistant, par exemple, à réduire la redondance des informations demandées aux entreprises et aux particuliers, dans un souci de simplification administrative, optimiser et à massifier les flux d'information vers la banque du sous-sol afin d'améliorer la connaissance des ressources disponibles. Il a par ailleurs pour objet de compléter l'habilitation afin de préciser le cadre juridique s'appliquant à la recherche et à l'exploitation des substances de carrières et de mines dans les fonds marins du domaine public.

lancement de grands projets miniers. Le présent amendement a donc pour objet de clarifier l'obligation de consultation publique des collectivités territoriales et des populations concernées en matière minière, à toutes les étapes

en remplaçant les mots « renforçant les modalités d'information et de participation des collectivités territoriales et du public » par les mots « mettant en place les modalités de consultation publique et obligatoire

toute son importance au stockage massif et intersaisonnier de l'hydrogène et prévoit de faciliter la réutilisation de cavités salines comme solution de stockage et de déstockage de l'électricité renouvelable. Il convient de rappeler qu'actuellement aucun site de stockage souterrain d'hydrogène n'existe en France, métropole comme en outre-mer. Ainsi, pour un projet relatif à l'exploitation d'un site de stockage d'hydrogène, l'exploitant devrait obtenir un permis exclusif une autorisation d'ouverture des travaux miniers une concession de stockage souterrain, pour un délai d'instruction pouvant être compris entre quatre et six ans. Néanmoins, de nombreux sites de cavités salines ou sont aujourd'hui répertoriés comme techniquement susceptibles d'accueillir un site de stockage d'hydrogène, notamment en reconversion de sites existants de stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures ou de produits chimiques. Ainsi convient-il d'habiliter le Gouvernement à envisager un cadre réglementaire spécifique pour le stockage souterrain de l'hydrogène, afin de raccourcir ces délais d'autorisation, pour des cavités salines déjà

d'hydrogène. Une ordonnance du 17 février 2021 relative à l'hydrogène permet déjà l'extension des titres d'exploitation de stockage souterrain de gaz combustible ou de gaz naturel en cours de validité à l'hydrogène. Toutefois, en l'absence de titre d'exploitation en cours de validité, la reconversion de sites en stockage souterrain d'hydrogène ne peut être envisagée que par une demande d'octroi d'un titre d'exploration. Si les travaux ont fait la preuve que le stockage d'hydrogène est réalisable, le titulaire du titre d'exploration pourra déposer une demande d'octroi d'un titre d'exploitation. Il est nécessaire d'appliquer à cette activité le cadre juridique protecteur du régime légal des stockages souterrains dès lors qu'elle comporte des enjeux environnementaux et de sécurité bien particuliers. Il ne me paraît donc pas souhaitable

Le texte adopté par la commission couvre l'essentiel de ces travaux en précisant que les dispositions à prendre par ordonnances devront « faciliter l'octroi de titres miniers pour la reconversion de sites d'extraction en sites de stockage, dans le respect des dispositions applicables aux stockages d'énergie calorifique introduites par l'article 45 de la loi [dite cette loi ne modifie que le code minier, si bien que ses dispositions transitoires, en l'occurrence son II, n'ont vocation à s'appliquer qu'à l'égard de dispositions du code minier. Ne sont donc pas concernées les dispositions relatives aux stockages souterrains contenues dans le code de l'environnement. Il en résulte un « angle mort », objet du présent amendement. Cet amendement vise exclusivement à combler ce « vide juridique

en prenant en compte la nécessité de conserver la notion de juste indemnisation du propriétaire des terrains situés au-dessus de la future mine au regard des contraintes engendrées par cette privation de la propriété du sous-sol ». Il s'agirait de faire un pas

Le montant de cette redevance tréfoncière payable en une fois est effectivement, monsieur Jacquin, de 15 euros par hectare, mais- attention -n'oublions pas que l'octroi d'une concession définit un périmètre

bien que son rendement reste extrêmement faible. J'émets donc un avis de sagesse sur cet amendement.

en Guyane, comme le réclament de nombreuses associations du territoire.

sous des maisons ou des lieux d'habitation, donner aux propriétaires réunis en association en application de l'article L. 154-1. Or, dans les faits, l'application de ces deux articles ne fonctionne pas.

L'adoption de cet amendement permettrait l'évaluation de l'application de cette disposition du code minier un rapport publié avant la rédaction de l'ordonnance portant sur les garanties financières. Cet amendement nous a été suggéré par l'association SEL'idaire, collectif de défense des propriétaires concernés par l'exploitation minière

La fin progressive des aides publiques directes ou indirectes aux combustibles fossiles est l'une des recommandations émises par la Commission européenne à l'attention de la France concernant son projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat. La France est aujourd'hui le deuxième exportateur mondial d'équipements et de services à l'industrie des hydrocarbures ; ce secteur réalise à l'étranger près de 70 % de son chiffre d'affaires.

ayant pour objet l'exploration ou l'exploitation de gisements d'hydrocarbures liquides dans le cadre de permis correspondant à des gisements non encore exploités à compter du 1 janvier 2025, ainsi que de ne plus accorder cette garantie

Cet amendement vise à obliger les établissements de crédit et les sociétés de gestion de portefeuille à mesurer les émissions de gaz à effet de serre dont sont responsables leurs investissements dans les entreprises se livrant à des activités d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures et de charbon,

les banques françaises ont financé les énergies fossiles pour 295 milliards de dollars depuis la signature de l'accord. Encore plus surprenant,

Face à cette contradiction, nous souhaitons rappeler que la transition écologique ne pourra s'opérer par la seule bonne volonté affichée des principaux acteurs financiers. Par sa permissivité, le cadre réglementaire actuel, qui

Dans le cadre de la loi de 2019 relative à l'énergie et au climat, c'est la commission des affaires économiques du Sénat qui a fait adopter le principe selon lequel les sociétés de gestion de portefeuille conçoivent et rendent publique une information sur les risques liés au changement climatique et à la biodiversité. et à la biodiversité. Elles doivent y retracer toute leur stratégie d'investissement, les moyens pour y parvenir, les critères et les méthodologies, ainsi que les droits de vote. Doivent notamment y figurer les investissements de ces sociétés qui contribuent à l'atteinte de nos engagements climatiques. Par ailleurs, le dispositif va bien plus loin que les seules sociétés de gestion puisque sont également visés les organismes mutualistes ou de sécurité sociale. Demande de retrait, sinon avis défavorable.

et de son décret d'application, paru récemment, ainsi que du droit européen, la part de leur encours alignée sur les énergies fossiles. Cet amendement doublonne donc des exigences qui sont déjà prévues par le droit. Ces mêmes acteurs de marché devront publier également d'importantes informations relatives à leur stratégie d'alignement sur les objectifs de température de l'accord de Paris : la mesure de l'exposition de leur portefeuille, la manière dont leur politique d'engagement et de vote répond à ces objectifs, ainsi que les mesures correctrices mises en place. De telles exigences viennent compléter un droit européen en cours de développement,

C'est donc tout un cadre de recevabilité qui est en train de se mettre en place aux niveaux national et européen afin que les acteurs du marché français se désengagent des énergies fossiles, tout en accompagnant la transition énergétique en conformité avec les objectifs de l'accord de Paris.

compter du 1 janvier 2022 les entreprises financières réduisent « progressivement la part de leurs actifs détenus dans les entreprises se livrant à des activités d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures et du charbon

Aujourd'hui, leur avis n'est plus que consultatif. Cela n'est pas acceptable, car ils sont aménageurs du territoire et doivent avoir un rôle décisionnel sur tout projet de construction : ils doivent définir des conditions d'installation acceptables pour les citoyens et positives pour le territoire. La parole

L'objet de cet amendement est de renforcer le rôle des élus locaux et des populations dans tous les projets éoliens, en convergence avec ce que vient de rappeler notre collègue Catherine Di Folco. Il faut bien reconnaître que, durant ces dernières années, voire ces dernières semaines encore, la multiplication de ces installations d'électricité a posé de sérieux problèmes. Cela engendre d'ailleurs parfois des conflits et des incompréhensions. Or la qualité des implantations dépend de la qualité de la concertation et de l'acceptation par les populations et les élus des projets en question. L'objectif, encore une fois, est de renforcer le rôle des élus locaux dans l'implantation des éoliennes afin de rendre leur avis plus déterminant quand il s'agit d'opérer de tels choix. Quel

à instituer un droit de veto de la commune pour l'ensemble des projets, et pas uniquement pour ceux soumis à une enquête publique. L'amendement n° 860 rectifié me semble satisfaire l'objectif porté par ces amendements identiques

j'insiste bien sur ce point - d'évolution du mix électrique et de développement de l'électricité en France, car nous avons des besoins,

faut également tenir compte des éléments de patrimoine remarquables que nous souhaitons préserver. Bref, tous ces points vont permettre d'établir une cartographie assez précise, qui sera une aide à la décision pour tout un chacun.

que va retomber une Bible ! Il faut donc bien, à un moment, fixer une méthode pour que nous puissions respecter nos propres engagements. Cela permettra également à chaque région de prendre sa part à l'effort collectif. C'est une programmation qui concerne notre pays tout entier, il n'y a pas de raison que certaines régions fassent une grosse part de l'effort et d'autres moins. Il est normal qu'il y ait une répartition. Une fois que nous disposerons de cette cartographie et que nous connaîtrons les objectifs région par région, il sera plus facile de déterminer,

investissent dans l'éolienne située près de chez eux et perçoivent des revenus quand celle-ci fonctionne. C'est plus intéressant que le livret A

... Le Sénat, longtemps considéré comme quelque peu jacobin, porteur d'une vision pompidolienne de la France et de la planification, est tout d'un coup saisi d'une frénésie de municipalisme libertaire ! C'est assez nouveau,

un village avec des mâts éoliens de 60 à 140 mètres de hauteur contre l'avis d'un conseil municipal ? À côté de cela, les services de l'État font démonter une fenêtre en PVC dans une zone classée ABF,

L'énergie éolienne, comme toute énergie, n'a pas tous les atouts. Il n'existe pas d'énergie propre, sans aucun impact. Nous sommes face à un principe de responsabilité : quelle est l'énergie qui nous apportera des bénéfices à court terme à court terme sans impact pour les générations futures ? Une éolienne rachète son énergie grise en huit mois, aucune autre source d'énergie, aucune autre technologie, n'en fait autant, il faut le rappeler ! Tout à coup, nous assistons à une campagne de dénigrement assez incroyable contre les éoliennes. On se pose tout un tas de questions qu'on ne s'est jamais posées pour aucune autre installation ou infrastructure. On entend parler du béton.

présentés, c'est sans doute que nous avons eu un effet de balancier beaucoup trop important, avec un développement anarchique des éoliennes, sans aucune concertation et sans que les élus locaux puissent dire leur mot sur les implantations potentielles. Je rappelle simplement à mes collègues

qu'il suffisait de faire des appels à manifestation d'intérêt (AMI) pour régler le problème de l'énergie dans notre pays était une lourde erreur.

L'objectif est de mieux établir la concertation et la consultation. Premièrement, avant le dépôt de l'autorisation environnementale, le dossier doit être remis à la commune d'implantation et à son maire.

Et la cohérence, c'est de donner le pouvoir au conseil municipal. qui sont souvent démunis face à l'implantation de parcs éoliens sur leur territoire, malgré le rôle fondamental qu'ils jouent en matière d'aménagement. Les maires réclament davantage de visibilité, mais aussi la possibilité de jouer un rôle décisif dans ces projets d'implantation. Je note que, s'agissant de l'information des communes concernées, un régime est déjà prévu à l'article L. 181-28-2 du code de l'environnement, lequel a d'ailleurs été introduit au Sénat par un amendement au projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique, dite loi ASAP, en 2020. Le périmètre n'est toutefois pas tout à fait identique à celui qui est préconisé dans l'amendement, puisque l'article que je viens de citer prévoit une information de l'ensemble des communes limitrophes. Nous pourrions retravailler la rédaction en commission mixte paritaire, afin de clarifier le régime d'information des communes.

baisser la part du nucléaire et trouver des substituts. « Le premier substitut au nucléaire, c'est la maîtrise de la consommation, grâce à l'efficacité énergétique croissante. Mais attention, au global la consommation d'électricité va augmenter car nous devons décarboner le transport et le chauffage.

l'hydrolien également, et on ne disposera pas d'assez de gaz vert pour décarboner le gaz et produire de l'électricité. Il nous faut donc faire du solaire et de l'éolien. Le solaire est bon marché, mais prend beaucoup de place : pour construire l'équivalent d'un réacteur nucléaire EPR, il faudrait disposer des panneaux photovoltaïques sur l'équivalent de 7 500 terrains de football Nous allons continuer à chercher de l'espace et poursuivre la recherche pour augmenter la productivité, mais le solaire seul ne suffira pas. Il nous faut donc absolument développer l'éolien. « La France a cinq fois moins d'éoliennes au kilomètre carré que l'Allemagne,

on ne pourra pas réussir la transition énergétique et le développement de la mobilité électrique sans l'éolien terrestre. Ce n'est pas possible, comme le montrent les scénarios de RTE présentés la semaine dernière.

monsieur le président, et que vous nous avez invités à la sobriété en termes de prise de parole, mais

de travailler plus sereinement.

lesquelles ont été supprimées par la loi du 15 avril 2013, dite loi Brottes. Cet outil permettait aux collectivités